certaines situations. Il tend à prévoir qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions permettant à un étudiant en santé de changer d'université entre le premier et le deuxième cycle, ainsi que les conditions dans lesquelles certains étudiants justifiant de certains grades, titres ou diplômes, notamment européens, pourront être admis directement en deuxième cycle.

Pour les autres candidats n'ayant pas bénéficié de cette dispense, des compétences complémentaires devront être évaluées au cours d'épreuves, notamment orales. Ces modalités d'admission favoriseraient la diversité des recrutements, tout en simplifiant la procédure.

d'autant que les universités feront sans doute face à d'importants problèmes de moyens pour déployer la réforme du premier cycle, ne serait-ce que pour l'organisation des épreuves orales. Je m'interroge cependant, monsieur Amiel, sur la compatibilité de votre proposition avec les objectifs affichés par le Gouvernement.

d'autres compétences. Il semble que les meilleurs candidats issus de filières différentes puissent être reconnus sur la base de critères d'excellence et qu'ils

Laurence Cohen, pour explication de vote.

Cet amendement vise à faire figurer, parmi les critères de sélection retenus pour accéder en deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, le projet professionnel d'un étudiant s'engageant à exercer en zone sous-dense. Il s'agit ainsi de valoriser le projet professionnel des étudiants qui s'engagent à travailler dans les zones à faible densité, comme cela se pratique en Australie, au Canada, au Japon et même dans certains États américains.

513 rectifié vise à permettre la prise en compte d'un projet d'installation en zone sous-dotée dans les modalités d'évaluation des étudiants en premier cycle et les conditions de délivrance des diplômes. également à permettre la prise en compte des projets professionnels d'installation en zone sous-dotée pour l'admission en deuxième cycle, qui serait alors facilitée.

que nous assignons aux études de santé. Je considère que leur premier objectif, et à dire vrai, à mon avis, leur seul véritable objectif, est de former les professionnels qui prendront demain les patients en charge. Il ne s'agit donc pas de répondre aux carences territoriales de l'offre de soins.

Implicitement, cela signifierait que ces zones devraient se contenter des professionnels qui ne seraient peut-être pas les meilleurs, mais qui seraient prêts à s'y installer et à y exercer. Par ailleurs, il existe déjà des outils visant à inciter les étudiants à envisager un exercice en zone sous-dotée. Je pense au CESP, le contrat d'engagement de service public, qui monte en puissance et qui n'est pas corrélé, lui, aux résultats universitaires. Cela me paraît beaucoup plus sain.

que le décret devra préciser concrètement la manière de parvenir à la diversification des profils universitaires en formation médicale, ce qui constitue l'un des objectifs centraux de la réforme. Cet amendement vise un pourcentage rigide d'étudiants qui devraient provenir de telle ou telle filière, ce qui pourrait être inadapté à la situation de certaines universités, mais à prévoir un pourcentage plafond d'étudiants provenant d'une même voie. Il me semble que ce serait un moyen efficace de ne pas recréer une nouvelle voie royale vers les études de santé, c'est-à-dire une sorte de Paces, et d'encourager les étudiants à s'inscrire dans d'autres parcours universitaires. Il me paraîtrait par ailleurs souhaitable que le décret laisse une certaine marge aux universités pour adapter l'objectif de diversification des profils à leur maquette de formation.

Néanmoins, il nous semble que les solutions proposées par les universités seront multiples. Fixer dans la loi des pourcentages nous paraît donc dangereux.

cette condition fait déjà partie de la formulation retenue par l'alinéa 9, qui vise les diplômes en santé validés à l'étranger « permettant d'exercer dans le pays de délivrance

parole est à M. Daniel Chasseing. La formation pratique des étudiants doit s'ouvrir à l'ensemble des structures agréées pour la formation ou auprès des maîtres de stage pour la formation des études de médecine, afin que les étudiants puissent découvrir les différentes modalités de l'exercice de la profession de médecin. Il convient aussi de proposer une professionnalisation précoce de la formation. En outre, la mise en contact des futurs médecins avec des réalités différentes de celles qu'ils rencontrent dans les hôpitaux périphériques complétera utilement leur formation. Quel est l'avis de la commission ? Les membres de

Par ailleurs, dans la mesure où, selon un rapport de l'IGAS de décembre 2017, les stages extrahospitaliers sont encore très peu répandus et où leur déploiement nécessitera l'agrément de nombreux maîtres de stage, il me paraîtrait assez peu sage de prévoir leur généralisation immédiate et obligatoire pour l'ensemble des études de médecine. Je pense enfin qu'il serait très difficile de mettre en place des stages ambulatoires en premier cycle. La réforme des études de santé suppose en effet que ce dernier soit un cycle d'orientation universitaire, afin de garantir l'intégration d'étudiants de différentes filières.

sur l'article. Nous avons unanimement regretté le manque de clarté de cet article réformant les modalités d'accès au troisième cycle des études médicales. Nous avons bien compris que les épreuves classantes nationales seraient supprimées. comme l'indique Alain Milon dans son rapport, la seule lecture de cet article, « même combinée à celle de l'étude d'impact, ne permet en effet pas de déterminer clairement les modalités futures d'affectation des étudiants par spécialité ». Nous déplorons donc une nouvelle fois le fait que tout ou presque soit renvoyé à un décret. Pourtant, nous partageons le constat selon lequel il était nécessaire de revoir ces ECN, qui occupaient une place trop importante dans les études de médecine et qui, comme pour les QCM de la Paces, ne prenaient pas assez en compte, par exemple, le projet professionnel ou encore les aptitudes des étudiants pour telle ou telle spécialité. Madame la ministre, nous espérons que vous allez pouvoir éclairer la représentation nationale, ainsi que les étudiants concernés, sur les modalités d'organisation de ce troisième cycle,

vers une spécialité. Le fait de conditionner l'orientation professionnelle des étudiants au rang de classement aux ECN a eu des effets délétères. J'en mentionnerai un qu'il me semble primordial de corriger : celui des représentations et des schémas que les étudiants intègrent au cours de leurs études et qui jouent un rôle déterminant dans l'orientation globale du système de santé. Il est ainsi absolument essentiel que l'évolution des formations et des cadres d'exercice des étudiants aille vers davantage de pluridisciplinarité, d'apprentissage des complémentarités et d'articulation entre les différentes compétences, afin de préparer à la diversité des rôles et des missions attendues. Car nos besoins de coordination des professionnels et les difficultés éprouvées à mettre en oeuvre cette coordination résultent aussi d'un défaut de polyvalence et d'expertise transversale acquis pendant les études. C'est en sortant du modèle de filiarisation et de surspécialisation que s'opérera la mue culturelle dont notre système de santé a tant besoin.

C'est pour aller dans ce sens que nous proposons de conditionner l'entrée en troisième cycle à la réalisation d'au moins un stage dans une zone sous-dotée. Nous discuterons également d'un dispositif travaillé avec la majorité sénatoriale et qui vise à faire de la dernière année du troisième cycle une année d'exercice en médecine ambulatoire, sous le statut de médecin adjoint. Ce dispositif soulagerait rapidement les territoires et serait à même, me semble-t-il, de recueillir l'assentiment des différentes travées de notre assemblée. La parole est à M. Stéphane Piednoir,

de leur formation, des étudiants sont sujets à des violences et des comportements qui n'ont pas leur place dans les universités et les centres hospitaliers universitaires, ni ailleurs, bien Les enquêtes sur les violences dans le milieu médical, notamment à l'encontre des étudiants, montrent des choses assez révoltantes. Une enquête de l'intersyndicale nationale des internes de 2017 fait apparaître que 9 % des internes ont subi une forme de harcèlement sexuel et que 47 % d'entre eux se disent victimes de sexisme au quotidien. Une autre enquête menée par deux doctorantes en médecine nous indique que près de 30 % des externes ont subi des violences sexuelles dans le cadre de leurs études. En mars 2018, la ministre de l'enseignement supérieur a annoncé des mesures contre les violences sexistes et sexuelles, notamment la mise en place d'une cellule d'accueil et d'écoute et le lancement d'une campagne de sensibilisation. en l'absence de procédure claire, notamment lorsque ces faits se déroulent dans le cadre des stages en santé, et en raison d'un fort sentiment d'impunité, on constate un très faible recours aux procédures disciplinaires.

Pour briser l'omerta et responsabiliser les acteurs, notamment au sein des CHU, il me paraîtrait important de modifier cette organisation et éventuellement de créer une instance disciplinaire à l'échelon du centre hospitalier et universitaire. J'avais déposé un amendement en ce sens,

C'est vers eux que nous nous tournons en toute confiance quand nous sommes souffrants. Nous leur confions notre santé, en espérant qu'ils seront en mesure de nous prescrire les traitements les plus appropriés, les plus efficaces et les moins coûteux. Selon le Dr Jacques Boulet, généraliste depuis vingt ans et directeur du Centre d'enseignement et de développement de l'homéopathie, l'homéopathie est un complément à la médecine classique, une possibilité thérapeutique supplémentaire. Nous considérons que l'homéopathie permet de soigner le patient, dont le bien-être est au centre de nos préoccupations, et de l'accompagner, souvent à travers un traitement préventif. Bien sûr, s'il est efficace, il est plus difficile à évaluer, puisque l'on ne tombe pas malade et que l'on n'a pas besoin d'un traitement allopathique plus fort. Selon les sondages, un médecin généraliste sur trois prescrit quotidiennement des médicaments homéopathiques. Les sages-femmes sont 78 % à les prescrire régulièrement et 100 % des pharmacies les intègrent dans leur pratique quotidienne. Cette méthode apporte une réponse adaptée et efficace dans 80 % des cas, notamment en ORL, en dermatologie, dans le traitement du stress, des insomnies et de la fatigue. Cela est vertueux et doit se poursuivre. Une longue histoire lie désormais nos concitoyennes et concitoyens au traitement homéopathique. J'ai moi-même été interpellée sur le sujet, et j'ai entendu les inquiétudes des patients particulièrement attachés à cette médecine qui leur donne entière satisfaction. Les médecins doivent pouvoir continuer à avoir le choix de prescrire en toute connaissance de cause de l'homéopathie, afin d'apporter aux patients confort et efficacité sur la durée. Si la polémique est vive autour du remboursement des médicaments homéopathiques en ce moment, nous maintenons que nos praticiens doivent être formés et à même de répondre à cet engouement et à la demande forte d'une médecine plus naturelle et plus douce, tout en prenant en compte les potentielles interactions avec les traitements déjà prescrits. La parole

l'on forme davantage des praticiens hospitaliers que des médecins, de nombreux étudiants en médecine arrivant à la fin de leur cycle de formation sans jamais être sortis de l'hôpital. Le président du conseil de l'ordre des médecins reconnaît lui-même que

organise une refonte des modalités d'accès au troisième cycle des études médicales, selon un mécanisme à trois étages comprenant la validation du deuxième cycle par l'obtention d'une note minimale, un nouvel examen des connaissances et des compétences ainsi qu'une personnalisation du parcours et des aspirations de l'étudiant dans le choix de sa spécialité. Il est très important que l'on puisse accéder aux soins de premier recours en milieu rural et périurbain.

Le troisième cycle des études de médecine permet aux étudiants qui ont validé leur deuxième cycle de se présenter aux épreuves classantes nationales et d'acquérir une spécialisation.

Les nouveaux examens comprendront trois parties qui nous paraissent essentielles : un contrôle des connaissances et des compétences médicales de base, à travers

nos collègues, qu'ils siègent dans des instances nationales particulières ou dans des commissions disciplinaires locales, ne sont ni formés ni équipés administrativement et juridiquement pour gérer ce genre de situations.

d'une réflexion sur un observatoire et un service d'accueil spécifiquement destinés aux internes, aux stagiaires et aux étudiants en médecine,

que l'organisation de la formation est un vecteur reconnu par tous comme essentiel, non seulement dans le projet professionnel d'installation des futurs médecins, mais également dans le choix de leur lieu d'implantation et de vie. C'est pourquoi nous vous proposons de reprendre une disposition adoptée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, puis supprimée en séance publique, qui conditionne l'accès à l'internat à la réalisation d'au moins un stage en zone sous-dotée en offre de soins ou caractérisée par des difficultés d'accès aux soins. Un praticien ne s'installant pas dans un milieu qu'il n'a jamais expérimenté, la réalisation de stages dans des environnements différents de ceux des centres urbains, en particulier dans les territoires périurbains ou ruraux, sera l'occasion de découvrir d'autres pratiques de la médecine et de donner l'envie de pratiquer dans ces territoires.

Pour autant, l'obligation posée par cet amendement nous apparaît trop contraignante à l'heure actuelle. Nous manquons de maîtres de stage en milieu libéral et, plus encore, en zones sous-dotées. Qui plus est, l'organisation de la formation universitaire ne permet pas aux étudiants de se déplacer raisonnablement du lieu où ils reçoivent leur cours à un lieu de stage si celui-ci est éloigné de l'université. Je me demande d'ailleurs si cela n'obligerait pas les pouvoirs publics à prendre en charge les solutions de transport, voire le logement de ces étudiants. Certes, il existe des zones sous-dotées facilement accessibles, mais ce n'est pas le cas de toutes ces zones. Cela créerait donc des distorsions d'équité entre les étudiants. Nous risquerions, en fin de compte, de faire redoubler des étudiants faute d'avoir pu leur proposer des stages correspondant à leur maquette obligatoire de formation.

Nous devons donc veiller à offrir à ces étudiants le meilleur cadre de formation ; cela me semble extrêmement important. Or envoyer des étudiants dans des zones qui manquent de maîtres de stage aboutirait à dégrader leur encadrement et donc leur formation. Gardons par ailleurs à l'esprit que les étudiants de deuxième cycle sont encore jeunes et dans l'incapacité de prendre en charge un patient. Si nous voulons que les stages en zones sous-denses aient une véritable utilité

Nous sommes tous d'accord pour dire que les représentations se forgent au cours du deuxième cycle, mais le passage à l'acte est compliqué ; il a toujours été compliqué. Ces représentations sont très anciennes ; si elles dataient du ministère de Marisol Touraine, ce serait simple

le CHU de Clermont-Ferrand a mis en place une politique en la matière et a même changé l'organisation pédagogique du trimestre afin que les étudiants puissent passer plusieurs semaines d'affilée en stage,

Guillotin, pour explication de vote.

Le scrutin est ouvert.

aurait pour avantage de faire découvrir la profession à l'étudiant tout en lui apportant une expérience utile. Aujourd'hui, un étudiant sur cinq ne découvre pas la médecine générale et effectue l'intégralité de son externat en centre hospitalier. Pour renforcer l'intérêt pour la médecine générale et lutter contre la désertification médicale, il est nécessaire de développer des stages en médecine générale dès le deuxième cycle des études médicales. L'attractivité de la profession pourra être renforcée par un accès généralisé à ces stages de deuxième cycle, ce qui n'est malheureusement pas acquis dans toutes les facultés, malgré l'obligation réglementaire. de la commission ? La commission est évidemment favorable à l'idée d'une généralisation des stages en milieu ambulatoire au sein du parcours des étudiants en médecine. La découverte de la médecine générale et de l'exercice libéral permet en effet, bien souvent, de susciter des vocations. Je crains toutefois qu'ériger à ce titre une obligation législative pour l'accès au troisième cycle ne pose des difficultés pour un certain nombre d'étudiants,

Nous devons donc nous montrer extrêmement prudents quant à l'inscription de telles obligations dans la loi. Mme la ministre pourra néanmoins nous apporter des précisions sur la manière dont la généralisation des stages en milieu ambulatoire au cours du deuxième cycle est envisagée par le Gouvernement, de manière très concrète. deux réserves relatives à la rédaction de cet amendement. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé dans son objet, son dispositif ne prévoit pas que ces stages de médecine générale devront avoir lieu en milieu ambulatoire ; les étudiants pourront satisfaire à l'obligation proposée dans les services hospitaliers de médecine générale.

de maîtres de stage agréés. Nous avons mobilisé les doyens et les départements de médecine générale pour identifier et former les maîtres de stage potentiels. C'est ce qui nous permet d'envisager aujourd'hui de tendre vers l'objectif

d'accès aux soins dans les territoires ruraux et dans certains quartiers des villes. Les difficultés d'accès aux soins sont au coeur du profond sentiment d'injustice et d'abandon ressenti par une grande majorité de nos concitoyens. Les médecins, les patients et les élus appellent, depuis plusieurs années, à des solutions structurantes qui répondraient enfin à l'urgence de la situation. Face à un problème complexe, mais pas insurmontable, et dont les causes sont multiples, nous pouvons faire plusieurs constats. seuls 12 % des jeunes diplômés décident de s'installer en milieu libéral à l'issue de leurs études. Ensuite, la mise en oeuvre d'un quelconque mécanisme de conventionnement sélectif reviendrait à grever la jeune génération de nouvelles obligations contraires à l'exercice d'une profession libérale ; elle pourrait décourager des vocations. Enfin, les mécanismes de régulation ont fait preuve de leur inefficacité partout où ils ont été mis en oeuvre. Par exemple, ce système a rapidement été abandonné en Allemagne, où les jeunes médecins ont soit refusé de se conventionner pour pouvoir s'installer librement, soit préféré se diriger vers les hôpitaux. Cela n'a fait qu'accentuer les différences territoriales. Un pari bien plus ambitieux serait celui de l'incitation et de l'accompagnement des jeunes professionnels dans les territoires, à travers une plus grande professionnalisation, principe fort qui serait inscrit dans la loi.

professionnel. Le même objectif serait atteint de la même façon pour un certain nombre de spécialités, telles que l'ophtalmologie. La dernière année du DES de médecine deviendrait ainsi une année professionnalisante hors hôpital, dans les territoires. Je me félicite de nouveau du travail constructif mené en commission des affaires sociales avec les différents groupes de cette assemblée.

Les étudiants en dernière année de troisième cycle de médecine générale pourraient être mis à disposition des hôpitaux de proximité pour intervenir en qualité de médecins adjoints dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. Cela permettrait de recourir à ces médecins adjoints lorsqu'une carence de premier recours est constatée par le conseil département de l'ordre, par le maire de la commune ou par la communauté professionnelle territoriale de santé. La dernière année deviendrait une année de professionnalisation hors hôpital, dans les territoires, sous la responsabilité d'un maître de stage, dans

Dans notre recherche et notre préoccupation, partagée évidemment sur toutes les travées de cette assemblée, je l'imagine, de proposer un dispositif efficient pour lutter contre les déserts médicaux, ou les zones sous-denses, le groupe socialiste a souhaité s'inscrire dans une démarche concertée, et ce dans un objectif d'intérêt général, pour répondre à ce qui est aujourd'hui une préoccupation de nos concitoyens. Nous tenons à remercier le président-rapporteur, Alain Milon, ainsi que nos collègues des autres groupes porteurs d'un amendement identique, d'avoir souscrit à cette démarche, qui, je pense, fait honneur à la Haute Assemblée.

était voté, une réponse efficace et rapide à la problématique des déserts médicaux, notamment en familiarisant les professionnels de santé

Je tiens à saluer les amendements identiques portés par nos collègues Corinne Imbert, Daniel Chasseing et Yves Daudigny, qui constituent un véritable élément de réponse aux difficultés que connaissent les zones sous-dotées. objet de prévoir que les étudiants de troisième cycle réalisent une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans ces zones. Une telle disposition permettrait notamment de lutter contre la désaffection pour l'exercice libéral des jeunes médecins. Le présent sous-amendement vise les mêmes objectifs en les confortant. Nous partons d'un constat simple, et mes collègues de l'Aveyron ou des Ardennes ne me contrediront pas : c'est parce que l'on connaît et que l'on apprécie un territoire que l'on se projette dans une installation. Ce n'est pas moi qui le dis ; ce sont les représentants des associations d'étudiants en médecine avec lesquels j'ai pu échanger au cours de mes auditions. La formation des médecins témoigne à l'heure actuelle d'un hospitalo-centrisme fort. Ainsi, alors qu'un stage obligatoire d'initiation à la médecine générale de trois mois est prévu pendant les études de médecine, nombreux sont les étudiants à ne pas l'effectuer. Pourtant, 83 % des étudiants qui l'ont réalisé ont indiqué qu'il leur avait donné envie de pratiquer la médecine générale. La Drees constatait néanmoins en 2017 que la médecine générale était la deuxième spécialité la moins attractive après la médecine du travail, alors même qu'elle fait défaut dans les zones sous-dotées. Dès lors, ce sous-amendement vise à préciser que, au moins une partie de l'année, la pratique ambulatoire en autonomie est réalisée en zone sous-dense. Il s'agit d'un dispositif relativement flexible dans la mesure où ce stage pourrait être réalisé dans le cadre d'un exercice partagé entre plusieurs structures ambulatoires. Nous proposons une mesure qui se veut pragmatique, tenant compte des nouveaux moyens déployés en faveur de l'accompagnement des futurs médecins dans la construction de leur projet professionnel. Ainsi, le nombre de médecins agréés maîtres de stage universitaires a augmenté de 14 % entre 2018 et 2019. Ils sont plus de 10 000 à ce jour. De surcroît, les internes qui choisissent d'effectuer un stage en zone sous-dense peuvent désormais bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide mensuelle de 200 euros. Ces nouveaux moyens doivent aller de pair avec une véritable impulsion politique visant à développer les stages dans ces zones sous-denses. L'objectif est que les jeunes puissent découvrir des territoires méconnus et envisager l'exercice d'une médecine plus polyvalente. Le sous-amendement

Toutes les analyses convergent : il est nécessaire, pour lutter contre les déserts médicaux, de faire connaître la pratique en cabinet libéral hors de l'hôpital public aux étudiants au travers de stages. L'amendement n° 1 rectifié, notamment, tend à répondre à cette demande. Dans toutes les lois récentes relatives à la santé, on retrouve cette incitation au stage chez des médecins de ville. En pratique, la très grande majorité des stages a lieu dans les CHU des grandes villes, où les étudiants poursuivent leurs études, parce que les CHU sont très demandeurs

Pourquoi la médecine générale serait-elle toujours en repli par rapport aux autres spécialités ? C'est une question que les enseignants en médecine générale, notamment,

après six années de premier et deuxième cycle, plus deux années de troisième cycle, le jeune médecin, plus que le vieil étudiant,

en pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones sous-denses, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire. Le sous-amendement n°

en pratique ambulatoire préprofessionnelle. Ils proposent d'atteindre cet objectif selon des modalités variables, mais proches dans l'esprit. La commission des affaires sociales a travaillé, je le répète, de façon transpartisane à la rédaction des amendements n 1 rectifié, 542 rectifié et présenter l'équilibre le plus satisfaisant. En premier lieu, les étudiants visés sont ceux de la dernière année du cursus médical, en médecine générale mais aussi dans d'autres spécialités qui seront précisées par décret. Cela permettra d'inclure certaines spécialités de premier recours, telles que l'ophtalmologie ou la gynécologie. En deuxième lieu, cette rédaction ne fait pas référence à des stages pratiques, ni simplement à une pratique hors CHU, mais bien à une pratique ambulatoire En troisième lieu, elle n'oblige pas les étudiants à trouver un lieu de pratique en zone sous-dotée, mais prévoit simplement que cette pratique sera faite en priorité dans ces zones, ce qui permettra d'éviter le redoublement d'étudiants qui n'auraient pas pu trouver de lieu de pratique. Enfin, elle ne précise pas le statut sous lequel interviendra cette pratique, celui de médecin adjoint, tel qu'il est prévu à l'article 5, nous ayant paru potentiellement limitatif.

aux sous-amendements n 419 rectifié et 826, car ils ne correspondent pas à l'équilibre transpartisan trouvé en commission. Nous considérons que l'ordre des médecins doit conserver un contrôle sur l'exercice des praticiens non inscrits au tableau de l'ordre. Nous considérons également que la priorité donnée à la pratique ambulatoire en zone sous-dotée

en pratique ambulatoire sous statut de médecin adjoint. Vous proposez, pour une liste de spécialités à définir- on comprend qu'il s'agira en priorité des spécialités de premier recours en plus de la médecine générale -, que la dernière année du que la dernière année du troisième cycle soit réalisée en pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones sous-denses. Pour la médecine générale, cela me paraît finalement assez cohérent avec ce qui est prévu dans le cadre du Saspas et de la phase de consolidation de la réforme du troisième cycle. Ainsi, nous proposons déjà que l'étudiant exerce en autonomie supervisée. L'objectif est bien d'accompagner l'étudiant en fin de cursus vers son autonomie complète d'exercice pour l'obtention de son DES. En dehors de la médecine générale, il n'est pas prévu à ce stade que cet exercice soit impérativement réalisé en ambulatoire, parce que cela nécessiterait de disposer, pour ces spécialités,

en établissement de santé. Certains parcours de formation le justifieront à l'évidence, et nous avons tout autant intérêt à favoriser également les stages dans les établissements hors CHU.

Le fait qu'une partie de la dernière année soit réalisée en zone sous-dense nous renvoie aux interrogations partagées précédemment sur le nombre de maîtres de stage, même si, ici, il ne s'agit pas d'accueillir les internes de la totalité des spécialités. Néanmoins, je suis

générale. Nous avons augmenté de 17 % le nombre de maîtres de stage universitaires entre 2017 et 2018. C'est une augmentation progressive, mais nous sommes encore loin de pouvoir accueillir la totalité des étudiants. Enfin, poser, comme vous le faites, le principe que cette dernière année soit réalisée sous statut de médecin adjoint ou en autonomie- ce que vous appelez professionnalisation avec l'implication dans le dispositif du conseil départemental de l'ordre des médecins et de l'URPS, nous éloigne à mon sens du processus de formation dans lequel cette dernière année s'inscrit, pour nous rapprocher d'un modèle qui s'apparente à ce que je qualifierai d'un quasi-exercice. Si je ne suis pas fermée à ce que les conditions d'exercice au cours de la dernière séquence de troisième cycle évoluent, de manière cohérente avec le processus d'autonomisation progressive que j'évoquais, il est impératif que cette dernière année

Ces amendements témoignent à l'évidence de la volonté de trouver un équilibre destiné à apporter de nouvelles réponses aux problématiques de l'accès aux soins, tout en tenant compte des contraintes fortes liées au processus de formation que nous avons rappelées,

supervisée, avec la certitude, donc, qu'un médecin généraliste supervise l'exercice de cette troisième et dernière année, même si l'étudiant gagne en autonomie. En outre, tous les amendements visant à rendre ces stages obligatoires me posent problème, parce qu'il faut pouvoir proposer une quantité de stages suffisante. Je souhaite continuer à prôner l'attractivité des territoires plutôt que

à ouvrir la possibilité qu'une partie des stages soit réalisée sous statut de médecin remplaçant ou adjoint. Nous nous éloignons là encore du processus de formation pour nous rapprocher d'un modèle de quasi-exercice. Je vous invite également à le retirer ; à défaut,

Les démarches transpartisanes ne sont pas si fréquentes, et, quand elles existent, nous sommes souvent au coeur d'enjeux d'intérêt général. C'est le cas ici. Je veux souligner l'équilibre de cette proposition, qui répond aux objectifs de formation des médecins, tout en visant l'intérêt général, dans des délais courts pour les populations des territoires, et tout en respectant le caractère libéral des professions concernées. Il n'y aura pas d'obligation d'installation à l'issue des stages de troisième année de troisième cycle, et la pratique ambulatoire en autonomie éclairera la prise de décision du médecin nouvellement diplômé, le moment venu, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

Nous n'avons pas le choix, il faut répondre à l'urgence, dans des territoires qui se sentent abandonnés ». Ces propos sont les vôtres, madame la ministre. Vous les avez tenus cet après-midi, voilà quelques heures. Je ne saurais mieux dire, sauf à ajouter que le moment est venu de leur donner un sens politique concret.

le Val-de-Marne, département d'Île-de-France, rien qu'aux urgences de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, il manque sept médecins. Je pourrais multiplier les exemples.

débat ! Si l'on s'en tient au dispositif existant et au contenu actuel du projet de loi, il n'y aura pas de résolution, dans un terme raisonnable, de la question de la désertification médicale. médicale. Les mesures incitatives sont utiles, mais elles mettent du temps à produire leurs effets, et ceux-ci sont insuffisants. Il faut imaginer un autre dispositif ! Ce qui me marque, dans la réponse de la ministre, comme dans les propos de Laurence Cohen, c'est un énorme non-dit. Actuellement, le troisième cycle dure trois ans, mais l'harmonisation européenne des cursus et l'arrêté d'avril 2017 prévoient que la phase de consolidation soit mise en oeuvre au 1 janvier 2020. Or personne ne nous en dit rien phase de consolidation, c'est la quatrième année du troisième cycle. L'harmonisation européenne prévoit même, éventuellement, une durée supérieure à une année. Il n'est en aucune manière question de prendre quelque moyen que ce soit aux hôpitaux. On ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il est question d'utiliser le temps médical supplémentaire de cette phase de consolidation pour le projeter là où tout le monde s'accorde à dire que le problème est le plus criant. Après, on se mettra bien d'accord, et la voie réglementaire sait être inventive, pour régler les questions. Ces amendements sont rédigés avec suffisamment

trois années dans le troisième cycle. Il faut passer à la quatrième année. Je ne comprends pas votre réaction, madame la ministre. Vous êtes allée à un congrès important ce week-end, comme vous nous l'avez dit, la presse spécialisée rapporte que vous aviez reconnu être favorable à ce que la dernière année du troisième cycle des internes de médecine générale se fasse en professionnalisation avec un statut de praticien adjoint. Oui ou non ? Si c'est non, dites-le-nous, mais si c'est oui, travaillons ensemble à cette solution ! En tout cas, si vous ne changez pas de position, vont arriver des mesures coercitives,

bref, car les collègues qui se sont exprimés avant moi l'ont fait de manière tout à fait remarquable et que je me reconnais totalement dans tout ce qui a été dit.

enfin, pour un grand nombre d'entre eux, ce qu'est l'exercice de la médecine en dehors d'un CHU. Si l'on veut avoir une petite chance qu'ils choisissent d'exercer leur profession

l'autre, que le troisième cycle de médecine générale en France durera non plus trois mais quatre années. C'est un amendement d'efficacité, dont les effets se

l'a indiqué ; à titre personnel, je ne suis pas favorable à ces propositions.

fait référence de nombreuses fois -, se fera en « pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ». Cela dit, c'est une responsabilité très importante, et, pour le Gouvernement,

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Mesdames les ministres, mes chers collègues, il est minuit passé. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l'examen de ce texte.

d'opacité en matière de processus de sélection des bacheliers et des bachelières. Au nom du secret des délibérations, la ministre avait considéré que le droit d'information des citoyens était caduc. Elle avait alors qu'aucun algorithme local n'avait été mis en place. Après avoir bataillé aux côtés des syndicalistes, universitaires et étudiants contre ces pratiques des universités, nous avons pu avoir confirmation de ce que nous dénoncions avec justesse.

dans son avis du 18 janvier 2019, en regrettant que la très grande majorité des universités ait refusé de communiquer les informations relatives à l'examen des dossiers de candidature.

ailleurs, le Défenseur des droits a pointé du doigt le secret des délibérations du jury, qui « ne doit pas s'opposer à l'information des candidats sur le contenu exact et la manière précise d'évaluation de leurs candidatures ». Il y a donc clairement eu de votre part, de votre part, madame la ministre, une première volonté de faire peser sur les épaules des établissements des pratiques que vos services ont encouragées, avant un rétropédalage visant à couvrir les universités. universités. Il me semble qu'appliquer le même dispositif aux études de médecine ne pourrait conduire qu'aux mêmes dérives. C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à rendre publique l'utilisation des algorithmes locaux dans le cadre des études de médecine. Quel

des processus de consultation et de concertation obligatoires, préalablement à la publication des textes réglementaires. Il n'est pas d'usage qu'un décret en Conseil d'État-

cursus permet en effet de former des cliniciens à la recherche fondamentale, clinique et translationnelle par l'acquisition d'une formation à la recherche et d'un doctorat de sciences, au cours des études de médecine. Grâce à cette double compétence, ils participent au développement des innovations cliniques, enjeu majeur pour les patients et la médecine française de demain. Le Gouvernement a indiqué vouloir prendre davantage en considération les à-côtés dans l'évolution des étudiants en médecine. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'inscrire directement dans la loi la prise en compte de ces doubles cursus, qui représentent une chance pour la France. Aujourd'hui, il paraît très difficile à un étudiant en médecine de poursuivre son cursus de sciences en raison des fortes exigences

Chantal Deseyne. Cet amendement vise à faire bénéficier les étudiants d'une formation mixte, hospitalière et libérale. Il me semble important que le décloisonnement intervienne dès les études médicales.